La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été dit. Tribune. Nous n'avons pas reçu. D'observation il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Notre ordre du jour appelle l'examen de la motion présentée. Par. Les présidents Patrick Kanner. La présidente, Éliane Assassi. Président Gontard. Et plusieurs de leurs collègues. Tendant proposer au président de la République de soumettre au référendum, le projet de loi de financement. Rectificatif. De la Sécurité sociale pour 2023. Je vais immédiatement donner la parole au président Kader, auteur de la motion. Monsieur le président. Allez-y,

monsieur le président. Monsieur le Ministre. Madame et monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, au nom de ma collègue Éliane Assassi présidente et de son groupe CRCE. au nom du président Guillaume Gontard. Et de son groupe geste et des élus de mon groupe SER. J'ai l'honneur de vous présenter cette motion tendant à proposer au président de la République de soumettre au référendum. Ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif pour 2023. 2023. FT moi de commencer par une citation. Toute la bataille menée depuis le XIXe siècle se trouve ainsi résumé. La bataille pour le temps de vivre. La conquête du temps de vie. Quelle était cette vie pour un prolétaire au 19ème siècle il n'y avait pas de retraite à la fin de la vie, il n'y avait pas de journée de repos. Il n'y avait pas de week-end. 42 ans plus tard, mes chers collègues. Ces mots du président François Mitterrand pendant sa campagne présidentielle de 81. Résonne avec force dans notre hémicycle. Il résonne aussi dans mon histoire personnelle. Moi enfant du Nord ce département où les gens ont 2 ans d'espérance de vie de moins que la moyenne nationale. Je sais ce que voulait dire le mot travail dans le bassin minier à Denain où doués dans les usines textiles de Lille, Roubaix ou Tourcoing ou dans l'industrie métallurgique à Maubeuge ou Dunkerque. Le combat de ma famille politique depuis le 1er jour a été de conquérir un peu de temps de vivre. Il a fallu toujours par tout temps sous tous les régimes politiques arraché aux puissants les concessions qu'il refusait. Aujourd'hui se tienne face à moi, ce qui veulent revenir sur ses conquêtes sociales toujours pour les mêmes raisons. L'argent, la rentabilité. Quoi qu'il en coûte, sur le plan social. Ce sont le président de la République. La Première ministre et son gouvernement, Monsieur le Ministre, les majorités de droite, qu'elle soit relative à l'Assemblée nationale ou indiscutable au Sénat. Ces forces ne sont pas simplement face à nous parlementaires de gauche cela n'aurait pas beaucoup d'importance. Elles sont face aux Français en opposition frontale. Aujourd'hui, nous nous battons pas pour leur arracher de nouvelles concessions. Nous aurions préféré finalement nous nous battons pour qu'il n'arrache pas du temps de vivre aux Français que pour des économies budgétaires. Ils ne mettent pas en place un nouvel impôt sur la vie. D'autres politiques bien plus solidaire sont possibles. Ils ont malheureusement choisi l'injustice plutôt que l'équité. La retraite par répartition. Mes chers collègues, est un des piliers de notre système de protection sociale. Ce sont les luttes sociales successives qui l'ont forgée les périodes historiques qui l'ont renforcé. On peut citer ici la libération et ces jours Jours heureux et 81 et ses grandes conquêtes sociales avec ce texte, vous ne vous attaquez pas seulement français, vous vous attaquez aussi un pan de notre histoire. Certes il n'y a rien d'étonnant à ce que la droite tente de détricoter notre modèle social. J'ai même chanson de commerce le gouvernement comme la majorité sénatoriale sont dans leur rôle. Le faire ainsi en revanche est inédit. Choisir une procédure parlementaire qui fait obstacle à la tenue d'un débat parlementaire serein éclairé et sincère pour une réforme d'une telle importance sans parler des risques d'inconstitutionnalité cet inédit fragiliser notre pays avec un texte qui semble avoir été griffonné sur un bout de table tant ses auteurs n'en maîtrise pas des contours exacts cet inédit faire émerger un front syndical uni, tant la concertation et raté sinon existantes. C'est inédit. Réussir à coaliser une écrasante majorité de Français, même parmi vos électeurs du 1er tour cet inédit. Je pourrais continuer comme cela longtemps. Revenons sur quelques points que je viens d'évoquer. Avant d'en détailler d'autres. Vous avez choisi de détourner l'objectif de l'article 47 1 de la Constitution pour contourner le Parlement. J'ai parlé hier de piraterie parlementaire je persiste et signe. Ses lois de financement au sein de notre constitution ne sont pas faites pour mettre en place une réforme de grande ampleur de notre système de retraites en dévoyant cette procédure. Vous aboutissait à un examen trop rapide et incomplet d'une réforme sociale importante qui relève de la loi ordinaire. Une réforme qui aurait dû d'ailleurs et ça a été dit hier, précédée d'une grande réflexion sur la place du travail dans notre société, la place des seniors l'égalité femmes-hommes en termes de salaire par exemple avec cette procédure. Ce texte pourrait potentiellement être promulgué sans aucun vote d'une des deux chambres. C'est un scandale, c'est un bras de fer que vous engagez avec les Français et leurs représentants. Mais vous ne trompez personne vous faites cela, Monsieur le Ministre, car vous n'avez pas de majorité parlementaire propres pour faire voter votre réforme. Par ailleurs, en utilisant cette procédure, vous prenez le risque que le Conseil constitutionnel censure les cavaliers sociaux comme vous a d'ailleurs prévenu le Conseil d'État. Si ce projet de loi est votée, il pourrait vous être reproché que ces dispositifs non pas un effet suffisamment directe sur les recettes ou les dépenses de la Sécurité sociale. Quand on enlèvera ses sucrettes. Il ne restera plus que la pilule amère. Outre les risques d'inconstitutionnalité que je viens d'évoquer le choix de ses modalités de débats abîme notre démocratie que l'on soit clair on empêchant le temps nécessaire à un débat de qualité. Le gouvernement et le 1er comptable de la dégradation du climat autour de ce débat parlementaire. L'obstruction. C'est d'abord vous les débarque tronqué, c'est d'abord vous le passage en force et d'abord vous. Ensuite. Avec ce texte. On ne sait pas si vous êtes coupable du prix ou d'incompétence temps vous avez varié dans vos explications. Cela fait plusieurs semaines que vous naviguez de contre-vérités en approximation. la retraite, la retraite des femmes sur les 1200 euros de pension minimale, vous semblez mal connaître votre texte et vous Découvrez ses effets négatifs au fur et à mesure de son examen surtout quand nos collègues députés vont aller chercher les informations à la source et vous voyez à quoi je peux faire allusion. S'ensuit une litanie de mensonges pour camoufler vos insuffisances et votre politique antisociale. Je ne m'attarde pas sur ces points ils seront largement débattues ces prochains jours. Mais s'attaquer avec autant de légèreté à la retraite par répartition est inacceptable, nous sommes face à un mécano bancals élaborés par des bricoleurs. Je l'ai dit, vous n'avez pas de majorité propre au Parlement pour faire cette réforme. La seule majorité, que vous avez, elle est contre vous, contre cette réforme, ce sont les Français. Le front syndical uni et il faut le souligner, a permis de faire émerger une mobilisation inédite pacifique. La plus forte depuis 30 ans le 7 mars prochain. Le monde du travail réaffirmera haut et fort dans la rue son opposition au report de l'âge légal de départ. Nous sommes aussi leur porte-voix et pour dire non à la retraite à 64 ans. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, écouter les Français. Ils ont un discours clair et Net de refus de votre réforme injuste. Entendez-vous aussi les paroles des salariés qui disent cette réforme, on ne peut pas on ne S'il s'oppose à ce point à votre projet, c'est qu'il perce à jour vos intentions profondes. Ils savent que vous êtes en train de faire des économies sur le dos des ouvriers, les employés qu'ils soient issus de la classe populaire comme de la classe moyenne. Cette obsession du moins d'impôts obsession du moins d'impôts de plus en plus dénoncées par les autorités de régulation financière. Vous voulez finalement la faire supporter à 6 Français actif sur 10, soit 18 millions de nos concitoyens sans aucun aucun effort demandé à cet extrême minorité de contribuables qui a tant bénéficié de l'hyper bouclier fiscal du président de la République depuis 2017. Ceux-là peuvent dormir en paix. Mes chers collègues. Emmanuel Macron veillent à leur intérêt. Les Français ont bien compris que le ruissellement c'était pour les autres. Le président de la République a été élu pour faire barrage à l'extrême droite. Les Français ne lui ont pas donné de majorité pour une telle régression sociale. C'est pour cette raison que vous ne pourrez pas faire passer cette réforme uniquement et autrement qu'en brutalisant la République avec cette réforme. Pour résumer, vous jouez avec le feu tant sur la forme que sur la, sur le fond et vous savez qui risque d'en profiter. Sur le plan politique. Nous appelons retrait de cette réforme, mes chers collègues. C'est clair et Net. Mais faute de retrait nous vous offrons une autre voie nous trois groupes de gauche vous offre une autre voie avec cette motion référendaire. Je demande au gouvernement de montrer son visage et d'assumer franchement sa politique face aux Français présenté leur le texte. Ils sont dans la rue, ils préféreraient aller sûrement aux urnes. Mon appel s'adresse aussi et la majorité sénatoriale qui a les moyens de voter cette motion fait honneur à votre famille politique au gaullisme. Vous qui chaque année répété que la réforme de notre système de retraite est indispensable pour que les Français continuent à avoir une retraite fait trancher cette question fondamentale par un référendum, comme le permet la Constitution imaginée par le général de Gaulle. Mai dernier mot monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mes derniers mots seront pour le président de la République lui-même. Ce président de la République qui a osé appeler il y a quelques jours au bon sens des Français pour défendre sa réforme. Le bon sens et de retirer cette réforme. À défaut, à défaut. À défaut d'avoir le courage de la présenter devant les Français. Mes chers collègues, au nom de nos 3 groupes et pour toutes ces raisons, j'encourage la haute assemblée a voté cette motion référendaire. Je vais donner la parole Je vais donner la parole à Madame la rapporteure générale de la commission des affaires sociales Madame Élisabeth Doineau. Madame Madame la rapporteure générale. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur. Le vice-président de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur de la branche vieillesse. Mes chers collègues. Monsieur le président, Kader, vous venez de présenter au nom de votre groupe et celui de la présidente, Éliane Assassi, et du président Guillaume Gontard, cette motion référendaire. Nous nous y attendions. Ce n'est pas une surprise. Vous dire si c'est une. Un outil. On ne va pas appeler ça une arme de destruction d'obstruction majeur. Sans doute pas sans doute pas. Chacun use us des outils qui là dans sa boîte à outils. je voudrais vous faire part de de de 2 éléments, d'abord une incompréhension et d'autre part une conviction. Pourquoi une incompréhension parce que Monsieur le Président. Je sais combien vous êtes attaché à la démocratie parlementaire vous avez tellement d'occasions de le montrer, vous avez tellement d'occasions de le prouver. Et là aujourd'hui vous nous proposez finalement un court-circuit on ne débattrait pas au Parlement on laisserait la rue choisir pour pour les Français. Alors je vois que ça vous fait réagir. C'est bien c'est bien, ça fait réagir ça fait ça fait réagir. Mais moi je voudrais vous rappeler monsieur Kanner les paroles de François Hollande. Qui était de gauche, il me semble et qui disait il faut respecter la démocratie représentative. Pourquoi élire des députés pourquoi élire des sénateurs si toutes les questions peuvent être posées au peuple français et celle François Hollande. Alors revenons à notre sujet si on posé la question aux Français vous voulez-vous de cette. Loi. Vous savez bien que c'est une question binaire, oui ou non répondre à une telle question évidemment demander des efforts aux Français, ils vont répondre non. Et d'ailleurs les sondages le montrent, mais si on leur dit vous voulez-vous sauver votre système de réforme par répartition, ils vous diront oui.

Ah ah. Il faut être attentif aux questions que l'on pose lors d'un référendum. Et en tout cas je ne pense pas qu'ici, ce soit une solution à adopter. Ma conviction, c'est que nous avons aujourd'hui un mur de dettes et ça c'est pas moi qui le dis, c'est encore un socialiste et Pierre Moscovici. Le président du Haut Conseil des finances publiques nous dit que nous avons un mur de dettes et que nous avons une montagne d'investissement une montagne d'investissement pour les armées pour le climat. Pour restaurer le service public. Bref, nous avons des investissements à faire 155 milliards de dettes encore à amortir sur la cadette. Vous imaginez un petit peu la somme que ça fait. Et donc moi je ne veux pas laisser cette décision, cette décision qui est lourde, j'en prends la responsabilité, je ne veux pas donner voilà au peuple français cette responsabilité parce que j'estime que nous avons à l'apprendre ici au Parlement. Je je voudrais, je voudrais aussi terminer.

je donne la parole au rapporteur de la branche vieillesse. De la commission des affaires sociales. Monsieur René-Paul Savary. Merci. Oui, effectivement on peut se poser la question référendaire. C'est tout à fait légitime, cela voudrait dire que l'on propose. Au peuple. Le texte sur lequel nous sommes amenés à délibérer. La démocratie est ainsi faite, donc nous refusons le débat. Nous proposons au peuple. Le texte de loi telle qu'il est ainsi formulée en conséquence. Ce n'est pas prendre en compte toutes les avancées de justice sociale que nous proposons c'est pas prendre en compte l'effort supplémentaire. Des mères de famille que nous. nous. Récompensant à travers une mesure tout à fait significative avec une pension meilleure ce n'est pas prendre en compte suffisamment l'usure professionnelle qui sera amélioré par rapport au texte dans ce que nous proposons c'est ne pas ça prend dans compte les avancées de justice en ce qui concerne une amélioration du dispositif de retraite progressive et en conséquence, c'est une question brute de décoffrage que vous refusez aujourd'hui de débattre. Deuxièmement, nous connaissons l'esprit des Français, toujours un peu franchouillard gaulois et qui ne répondent pas, qui ne répondent pas forcément directement à la question et le référendum et si sensible à la façon de poser la question. Si vous leur aviez posé la question. Quand vous avez fait la réforme Touraine. Pourquoi vous ne l'avez pas fait vous l'aurez rien demandé quoi que l'on travaille de 41 ans et demi à 43 ans parce que c'est ça la réalité. Vous leur rien demander quoi aux Français, aux jeunes de 16 ans, vous savez ce qu'ont quatre à cinq trimestres avant la fin de la ramener à votre loi à ces jeunes de 16 ans. Vous leur auriez proposé, êtes-vous d'accord de travailler 45 ans. Dans la loi là. On leur propose de travailler moins. Voilà la façon de poser la question et si demain vous leur dites. Et demain, vous leur dites. On a des difficultés, mais voyez-vous, on ne veut pas fait d'effort. Est ce que vous voulez travailler de 62 à se passer ce serait la façon dont vous poseriez la question, moi je la poserai pas. Comme ça je dirais écoutez si nous ne prenons pas nos responsabilités. Est ce que vous voulez que nos enfants travaillent 65 ans plutôt 64 ans et vous verrez que la réponse sera différente. Et si vous avez entendu. Si vous avez entendu différentes manifestations. Nous les avons entendus mais nous avons aussi écouter les syndicats. Que nous disent les syndicats. Que nous dit la CGT. Que nous dit la CFDT. Il faut débattre du texte. Il faut débattre du texte. J'ai été encore en discussion avec une déléguée CGT de mon département, elle m'a dit monsieur le sénateur, pour débattre du texte. Nous suivons les syndicats. Nous suivrons les syndicats. En conséquence, vous l'avez bien compris, je ne laisserai pas planer le suspense plus longtemps j'émets un avis défavorable. Ministre. La parole La parole est maintenant notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Merci beaucoup monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Madame la rapporteure générale monsieur le rapporteur. Chers collègues. Évidemment, les sénateurs ne peuvent pas se décharger de leur mission d'examen de débats de vote d'un tel projet de loi, ce serait. Purement et simplement démissionner et alors que le débat s'engage à peine vous proposez de l'interrompre. Ben en effet c'est l'article 68 de notre règlement en cas d'adoption de cette motion, que se passerait-il elle suspend les débats. Elle va à l'Assemblée nationale. Son sort est connue. Bref tout ça pour ça et je rappelle que le Sénat un rôle tout particulier en ce moment, celui de débattre des 20 articles du projet de loi parce que ce n'a pas pu être fait à l'Assemblée nationale où seulement deux des 20 articles ont été examinés. D'ailleurs, tant Philippe Martinez que Laurent Berger, le regretté. Je cite ce dernier qui dit qu'a parlé d'un spectacle indigne et honteux. Et donc ce souhait d'un débat au fond du texte. C'est pas une lubie, ni de la majorité présidentielle, ni de la majorité sénatoriale. C'est un devoir vis-à-vis des partenaires sociaux, c'est un devoir vis-à-vis des Français et hélas avec cette motion vous voulez et ce qui fait le débat preuve aussi on est le dépôt d'amendements par milliers parce que votre ligne elle est simple hein elle est pas bouger pas fâché, mais les Français vous dit aussi pas gouverné depuis 2 présidentielle et donc nous nous avons une conscience aiguë de la nécessité d'agir. Également une conviction que le Parlement peut être utile et donc nous ne pouvons accepter cette motion. D'ailleurs si je refais un peu le film des derniers débats. Que ne l'avez-vous utilisé. Écoutez les Français nous dit le président Kader mais moi je me souviens avec le président mi-longs en 2016 sur la loi travail qui mettait en place une véritable révolution copernicienne. Vous savez, grâce à la loi travail, on peut travailler 46 heures par semaine pendant 12 semaines. Est ce que vous voulez proposer au référendum. Non, 2 Français sur 3 à l'époque voulait le retrait de cette loi. Avez-vous fait un référendum à nouveau non. Et puis si on parle des retraites. La loi Touraine en 2014 elle augmenter la durée d'assurance à 43 ans. La présidente. Laurence Cohen à l'époque disait ça va frapper de plein fouet les femmes vous en faites aujourd'hui un choix de société. L'avez-vous soumis à référendum à l'époque non. Alors je reconnais la constance du groupe CRCE parce que le groupe CRCE déposer des motions porter le fer. Mais du côté des socialistes, on ne peut pas dire que il y a cette cohérence et cette constance et puis pardon mais si on parle de la retraite à 60 ans en 81. Elle a été instituée. Non pas par référendum, même pas par débat parlementaires par ordonnance. Le Parlement a été mis hors d'état de débattre à l'époque. Et à l'époque et à l'époque Robert Lion, directeur de cabinet du Premier ministre hein avertissait sur les risques d'une retraite à 60 ans. Dans son rapport vieillir demain je vous y renvoie. Et donc. On le voit, si référendum il y avait il faudrait également soumettre. Au choix des Français vos propositions. Je vois le succès qu'il y aurait, êtes-vous prêt à renoncer à 10% de vos pensions. Êtes-vous prêt à payer 15 milliards d'euros d'impôts supplémentaires chaque année. Et puis le référendum. Comment faites-vous pour. Recueillir l'assentiment de celles et de ceux pour qui nous faisons cette retraite, ceux qui ont cinq mois, ceux qui ont 5 ans ceux qui ont 10 ans ceux qui ont 15 ans qui ne peuvent pas glisser un bulletin de vote dans un dans une urne et qui pourtant ont le droit à une retraite. Et ils n'ont pas forcément droit justement un régime qui auraient failli par banqueroute. Alors que faire. Eh bien écoutez je me remémore les propos du questeur Alain Anziani. En réponse à une motion référendaire en 2010 dans cet hémicycle. Et que disait Alain Anziani il disait l'autre façon de consulter le peuple. Sur les retraites, c'est l'élection présidentielle, hé bien ça tombe bien, le président de la République dès avant le 1er tour, il a posé le sujet, il a dit ce qu'il allait faire le peuvent s'est exprimé au 1er tour, il a été clair, il l'a envoyé au second. Et puis, écoutez. Vous pouvez prendre le par tous les bouts, vos collègues. Socialistes ou sociaux-démocrates. Ailleurs en Europe. Ils n'ont pas fait la politique de l'autruche. Ils ont réformé dans le même sens que ce que nous proposons c'est le Portugal de José Socrates, 66 ans, c'est l'Espagne de José Luis Zapatero, 66 ans, c'est la Grèce d'Alexis Tsipras souvenez-vous Syriza Syriza, 67 ans. Alors oui il faut apporter des réponses pour les retraités d'aujourd'hui et de demain, et vite. Il y a urgence pour consolider le système urgence pour améliorer les droits urgence pour travailler sur ce projet de loi le groupe RDPI votera donc contre cette motion référendaire pour que nous puissions poursuivent l'examen du texte, faire notre travail de parlementaire au service des Français et c'est d'ailleurs tout le sens de cette belle analyse livrée dans pouvoir que je vous livre l'article 11 puisque cette ce celui-là dont il s'agit doit être utilisé avec précaution. À propos de texte peu nombreux et simples dans leur rédaction sinon il serait préférable que la population des Français fut éclairé par un large débat parlementaire. François Mitterrand, avril 1988. Alors je le dis à nos collègues de l'opposition soyez mitterrandien, soyez à la hauteur de votre héritage politique ne le reniez pas ce n'est pas une défroque un vêtements usagés éclairé. Donc les Français par ce large débat parlementaire et rejetons cette motion. Merci. Merci. Donner la parole à notre collègue Émilienne Pomerol pour le groupe socialiste. Écologiste et républicain. La parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Au lendemain de la victoire de 1945, le gouvernement proclame dans sa Constitution de 1946 au sein du préambule que la nation garantit à tous, notamment la enfant à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui en raison de son âge, son état physique ou mental. La situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Les forces vives de la résistance ont donc appliquer le programme des jours heureux et ainsi la France a bâti la sécurité sociale hésite un moment historique. Il traduit la solidarité en particulier, grâce à la création du système de retraite qui permet à chacun de bénéficier de droits acquis grâce à son travail pour profiter de la vie, c'est la solidarité intergénérationnelle. La politique c'est changer la vie. Changer la vie, ici et maintenant. C'était le thème que nous portions de nous, les socialistes en 1981. Et c'est ce que François Mitterrand grimper. Parmi les grandes avancées sociales, il a mis en place la retraite à 60 ans parce que nous savions et nous avons toujours combien le travail peut être pénible et endommagé la santé des gens, il n'y a qu'à voir 35 pour % des ouvriers aujourd'hui seulement travaillent au delà de 60 ans parce que leur santé ne leur permet pas d'aller au-delà. Or, ce gouvernement a lui a enlevé les critères de pénibilité. La politique du gouvernement actuel ces de dégrader la vie, notamment celle des femmes, des précaires, celle dont la carrière est longue. Changer la vie, c'est pour nous pour l'aide-soignante d'Aurillac. La femme de ménage de Saint-Denis ou encore la coiffeuse de mort là si cette France du travail qui crie sa colère dans ces cortèges dans tous les territoires. La retraite avait été pensé comme un nouveau salaire qui permet d'employés librement à son rythme dans des relations autre que des relations marchandes au bénéfice de la société toute entière. La France tire de ces retraités une richesse que des tableaux comptables ne peuvent faire faire ressortir. Ils sont ainsi le premier à être engagé dans notre tissu associatif, ils assurent des millions d'heures de garde d'enfants, ils sont les élus de nos communes. Vous avez donc réduire de deux ans leur engagement au bénéfice de la société, contrairement au gouvernement. Les Français connaissent cette richesse et demeurent attachés. Au système nazi Kurdi sociale et de retraite ces dernières semaines. Ils ont par million manifester leur rejet dans la rue et ont rejoint le front syndical uni qui s'est créé contre votre réforme par la faute du gouvernement et à cause de votre vision purement comptable, nous assistons ainsi aux plus grandes manifestations depuis 30 ans ensemble tous lutte pour empêcher votre réforme injuste brutale et inutile. Le 7 mars, les syndicats n'auront d'non le 8 mars, les femmes d'Iran. Non le 9 mars, les étudiants dire Iran non et enfin le 10 mars les marches pour le climat diront non à votre réforme. Injuste et libéral. Vous prenez le risque par votre dogmatisme de mettre le pays à l'arrêt. Alors dans un esprit de Concorde. Nous vous proposons une j'abattoirs le référendum si c'est là. Le référendum a été inscrit dans notre Constitution pour que les Français puissent décider par eux-mêmes de la voix, que les politiques doivent reprendre le général de Gaulle à part 4 fois décidé s'en remettre à Jess populaire les crises que la France travailler traversé d'alors ont amené nos concitoyens à prendre leurs responsabilités pour décider de leur avenir. Or, l'avenir des Français. C'est précisément l'enjeu de cette réforme, il est prioritaire d'intégrer le français dans la discussion et associer à la construction de leur future société aujourd'hui plus de 2 tiers des Français se pose à votre réforme des millions l'ont créé dans la rue et le gouvernement ne dispose pas de la légitimité pour faire cette réforme, contrairement à ce que dit le président de la République. Monsieur Macron. Il n'a pas été élu sur son programme mais pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et d'ailleurs le président de la République n'a pas obtenu de légitimité, puisque les législatives suivantes ne lui ont pas donné de majorité ce qui l'oblige à composer avec les élus de droite, la souveraineté nationale appartient au peuple. Ainsi, lorsque le peuple est en désaccord avec ses représentants. Il ne reste que la voie du référendum. Aujourd'hui, je sais qu'à ma gauche, le choix de poser la question à nos concitoyennes a été prise. Je me tourne alors vers ma droite par une curieuse coïncidence que seule l'histoire s'est créée il reviennent au peuple. Au groupe pardon héritée du gaullisme de trancher la question de proposer ou non un référendum. Mes chers collègues. Il vous appartient d'offrir à nouveau au peuple les clés de son destin. de son destin. Parole à notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, demander un référendum sur ce projet de recul de l'âge de départ à la retraite sonne aujourd'hui comme une évidence. Monsieur le Ministre, mes chers collègues de la majorité présidentielle et sénatoriales aujourd'hui main dans la main, je vous le redis, le rejet de cette mesure provocatrice et massif dans ce pays, c'est une provocation de répondre par l'obligation de travailler plus longtemps à la détresse à l'angoisse de la population frappée par la crise du Covid, victime d'une précarité croissante dans le travail et dans la vie quotidienne et qui subit une inflation à 2 chiffres sur les produits alimentaires et de première nécessité. C'est une provocation à l'égard des femmes déjà victimes de discrimination en matière salariale d'évolution de carrière plutôt que l'égalité, vous ajoutez de la maltraitance en rallongeant soit leur travail soit leur période de chômage, car vous savez bien qu'en reculant l'âge de la retraite, c'est le chômage des seniors que vous. Le message que vous envoyez aux femmes et des plus cyniques, vous leur dites qu'elles vont travailler plus longtemps mais que l'écart entre leur pension et celle des hommes qui s'élève, faut-il le rappeler à 40% va être moindres mais ce que veulent les femmes ce n'est pas un écart cosmétique, c'est l'égalité. Depuis 2017, le président Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale. Alors mettez en adéquation ses paroles et ses actes. L'égalité salariale et l'égalité d'accès à l'emploi des femmes permettrait de résoudre le pseudo déficit qui justifie votre réforme inique. Avec les amis de mon groupe mais aussi de toute la gauche sénatoriale. Nous sommes scandalisés par les propositions de monsieur Retailleau. S'appuyant sur une idéologie familialiste nationaliste du n'est pas que je n'ose rappeler non monsieur Retailleau. Les femmes ne peuvent avoir pour seule solution afin d'éviter de travailler jusqu'à un âge à déterminer que de faire plus d'enfants. Nous vous demandons de retirer cette proposition par dignité. C'est une provocation à l'égard de la jeunesse. Durement éprouvés par le Covid par un monde incertain des guerres dans de nombreux pays la menace d'une 3ème guerre mondiale une jeunesse confrontée à cet inquiétant réchauffement climatique soumis à un parcours scolaire et universitaire de plus en plus sélectifs dans des conditions de plus en plus difficile. Que proposez-vous à la jeunesse un service national universel autoritaire une forme d'embrigadement insupportable pour celles et ceux qui ont soif de liberté et une carrière qui ne ne se terminera qu'avec la vieillesse car quel étudiant pourra espérer une retraite avant 70 ans c'est une provocation pour les travailleuses et les travailleurs y compris celles et ceux qui exercent des métiers pénibles ont une carrière longue ou. Aujourd'hui, celles, ceux que vous qu'ouvriers hypocritement de louanges ces premières et premiers de corvée durant la crise du Covid. Oui, la colère est grande, et elle s'amplifie la mobilisation à compter du 7 mars s'annonce massive. C'est une très bonne nouvelle et hier dans l'hémicycle, nous avons pu vivre cette opposition entre 2 projets de société aux antipodes dans un clivage droite- gauche enfin assumer y compris Macron et son gouvernement veut passer aux forceps en utilisant cette procédure de l'article 47 hein si décrié depuis sa mise en oeuvre pour l'examen de cette réforme des retraites et qui relève du détournement de procédure, nous l'avons affirmé hier vous violer la Constitution pour imposer cette réforme vous contraignait le Parlement vous tentez de le soumettre et nous sommes choqués par cette majorité sénatoriale qui avait affiché son statut de contrepouvoir de lieux de résistance à l'autoritarisme de monsieur Macron à ce mépris du Parlement et qui aujourd'hui l'accompagne avec complaisance, mes chers collègues vous accompagner le président de la République dans cette mise au pas du Parlement, pire, cet engin aux mains du Parlement puisqu'un texte non soumis au vote de l'Assemblée nationale et peut être même non soumis au vote des 2 chambres. Si le gouvernement n'ouvrent pas plus de jours de débat, un débat et une adoption CMP dominé par des parlementaires LR pourtant en perte d'influence dans l'opinion publique. C'est un coup de force âge Titus Lionel il faut donner au peuple et moyen d'y résister, lui donner les moyens, c'est lui donner la parole c'est soumettre ce texte au référendum qui ici peut oser dire alors que plus de 90% des actifs rejette le texte, restons entre nous au Sénat valide ce texte fondamental dans un temps contraint et barrant la route à l'expression populaire tout vote contre cette motion référendaire est un acte grave contre la démocratie chez et ce qui sortait trop dans ce déni de démocratie porteront la responsabilité de la mise à l'arrêt du pays et d'une légitime révolte avec le groupe CRCE je vous appelle donc seuls aliments à voter cette motion référendaire sans hésiter. Il avait donné maintenant la parole à notre collègue Olivier Henno. Pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Mesdames, messieurs les rapporteurs chers collègues un 1er mot à nouveau pour saluer les rapporteurs leur travail. À la fois sur. Le fond du texte, mais aussi du point de vue de, de l'analyse. Et puis sur la méthode. Et saluer leur. Leur calme. Leur modération c'est important le calmer la modération hein, on vient de le voir a pas cité de d'écoute, de dialogue, d'échanges et de pédagogie et même leur sens de la formule, ils viennent d'en faire la démonstration, votre travail grandit notre institution le Sénat et donc merci nous sommes rassemblés ce matin pour discuter d'une motion référendaire. Je veux tout de suite au nom du groupe UC dire mais sans l'ombre d'une hésitation que nous ne la voterons pas pour des raisons d'opportunité mais également pour des raisons de fond, du point de vue de l'opportunité nous sommes rassemblés pour débattre de l'avenir de notre système de retraite et pour nous il serait tout à fait inopportun de refuser ce débat s'exonérer du débat sur les retraites, ici et maintenant. En choisissant le référendum. Cela reviendrait pour nous a refusé l'obstacle et ça c'est pas une méthode pour nous. Voilà pour l'opportunité, sur le fond, notre groupe j'ajoute appartient à une tradition politique qui pense que le référendum doit être réservé à la matière institutionnelle pour les questions sociétales, comme pour les questions économiques et sociales. Nous pensons que c'est le rôle du Parlement de débattre et de voter. J'ajoute que cette motion référendaire. La voter. Reviendrait à créer un redoutable. Précédent. Parce que ça nous interdirait pour longtemps de débattre des retraites ici au Parlement parce que pourquoi on fera un référendum maintenant et pas ensuite sur des débats comme ça et pourquoi sur des questions aussi essentielles que des questions sociétales, économiques et sociales on demanderait pas systématiquement à référendum et donc un précédent comme cela serait tout à fait irresponsable, ce serait d'ailleurs porté un bien mauvais coup à la démocratie parlementaire. Donc pour nous, c'est clairement non à cette motion référendaire je veux à présent profiter de temps qu'il me reste pour discuter du texte sur les retraites mais aussi du contexte de ce débat. Vous l'avez compris hier au travers des interventions de Hervé Marseille et de Jean Marie Lorraine Berg, notre groupe s'est clairement positionné pour cette réforme. Ah oui mais alors quand on dit oui mais quelques fois, c'est un petit oui il a un grand mais mais non là c'est une forme d'équilibre et c'est un oui mais mais c'est un oui bien sûr et hein mais parce qu'il faut améliorer ce texte. Ce sera d'ailleurs dans une double volonté, une, un certain équilibre bien sûr mais la volonté d'enrichir ce texte notamment sur les, pour les femmes les les familles les carrières longues. Et l'emploi des seniors, nous saluons et approuvons d'ailleurs les avancées de la commission. En termes d'équité en terme de justice mais nous proposerons aussi par l'intermédiaire de quelques amendements d'aller plus loin encore, tout en veillant à l'équilibre financier du texte est fondamental. Cette question de l'équilibre financier de cette réforme parce qu'il faut qu'elle vaille la peine, sinon les Français ne manquerait pas de nous dire ben tout ça pour ça et ils auraient raison, un système de retraite repose sur la solidarité entre les générations. Voilà pourquoi je ne comprends toujours pas la timidité du gouvernement en matière de politique familiale à l'aube de ce débat sur les retraites, le choix du gouvernement, lors du dernier PLFSS, il faut le rappeler d'avoir privé la branche famille de 2 milliards d'euros m'apparaît encore plus aujourd'hui totalement inapproprié. C'est pourquoi l'un de nos amendements phares sera celui qui prévoit une mesure d'âge ça va pas plaire sur certains mots tout simples à retraite à 60 ans pour les familles de 2 enfants et 64 ans pour les familles de 3 enfants et plus. Je ne crains pas d'assurer d'assumer. On est un certain nombre ici dans cet hémicycle. L'urgence d'une politique familiale et nataliste au moment où la France ne renouvellent plus les générations, avec un taux de natalité inférieurs à deux ça sonne comme une évidence. Bien sûr vous l'avez compris, notre groupe est très attachés à notre système de financement de retraites par répartition. C'est pourquoi nous voulons aborder ce débat les yeux ouverts et en toute lucidité, se donner les moyens de financer la retraite de plus de 20 millions de retraités, et non seulement à des films mais une exigence morale qui impose d'imposer d'anticiper les besoins de financement croissant. Nous partageons le principe que seul le travail, et je dirais même l'augmentation de la quantité de travail produite par notre pays peut garantir le financement de notre protection sociale et donc le financement de la branche vieillesse et des retraites mais au-delà de la question du financement, nous sommes attachés à la valeur travail, ce n'est pas sur les bancs du groupe UC que se fera entendre un éloge de la paresse. C'est pourquoi il nous semble indispensable d'organiser dans les meilleurs délais un débat sur le travail et la rémunération des salariés, j'ai la conviction que les partenaires sociaux sont prêts à aborder cette discussion en responsabilité. Un tel débat sur le travail nous permettra d'aborder dans la sérénité, je le répète cette question essentielle de l'emploi des seniors un index seniors est un 1er geste il est nécessaire, mais sera-t-il suffisant. J'ai bien peur que la réussite de cette réforme passe par la possibilité de tous et tous de s'épanouir dans son emploi, jusqu'à 64 ans d'ailleurs, pour nous, le débat sur le travail est indispensable pour preuve un sondage publié hier. Démontre combien les Françaises et les Français en viennent parfois à douter de l'importance du travail au lendemain de la crise Covid. Ah si je ne me résous pas à lire que 58% des Français contre 49 en 2019 voient le travail comme contrainte quand 42% seulement y voit un moyen de se réaliser. Ils étaient 51% en 2019 avoir un moyen de se réaliser, ce recul est alarmant pour notre pays. Je refuse de compter parmi les déclinistes. Mais reconnaissons que ce changement profond s'il venait à durer, s'il est anthropologique est un germe de déclin de notre pays. Ce débat sur le travail dans la société post-Covid doit permettre d'approfondir, de nouveau sujets je comprends je pense au travail de seniors, je, je le répète, à une augmentation des salaires. À la veille du retour de l'inflation, conséquence peu surprenante du poids qu'il en coûte et de l'injection massive d'argent public dans l'économie, je pense à la pénibilité des métiers, je pense à la question des métiers en tension, je pense enfin à la formation tout au long de la vie qui doit donner à celles et à ceux qui en ont la volonté de pouvoir changer de métier. Le bien-être au travail l'épanouissement au travail, voilà le défi auquel nous sommes collectivement confrontés même si nous pensons qu'il faut aller plus loin en terme d'équité, de justice, nous faisons le pari qu'il y aura une réforme des retraites. Mais au lendemain de l'adoption de cette réforme, il y aura obligation de recoudre notre tissu social et ce sera notre dernière remarque au nom du groupe UC comme l'a formulé hier notre président nous demandons l'organisation d'une conférence sociale qui pourrait avoir pour objectif la refondation du paritarisme pour recréer la confiance dans ce pays qui est dégradé, la rémunération des salariés et puis la place du travail dans nos vies, mais chers collègues, vous l'avez compris, notre groupe a envie de débattre, d'aller au bout de ce débat de conclure ce débat, c'est le rôle et la mission et la responsabilité du Sénat et donc pour toutes ces raisons que je viens d'énoncer notre groupe ne votera pas cette motion référendaire. Je vous remercie. Monsieur le président. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre. Mal président la commission des affaires sociales mesdames et messieurs les rapporteurs.

retiennent débat pour un groupe. La réponse est oui. Nous savons combien la constitution dans les moyens de faire passer un texte si le gouvernement est déterminé à le faire ah Restless. Hier après-midi par la double voix du ministre. Nous avons bien entendu que comme pour lui, il était souhaitable mais aussi que la réforme était incontournable. Les regards sont braqués sur le Sénat, Assemblée, bien sûr ça faut-il démontrer quel que soit le six qui voulait qu'on ne montre espérons qu'il soit au moins empreint de respect. Ce que nous avons pas eu à l'Assemblée nationale a choqué beaucoup de nos concitoyens. Beaucoup des groupes on ça nous de travailler à l'amour sur ce texte. Depuis des semaines pour tenter d'améliorer cette réforme des retraites au sein du RDSE. Non écoutez, syndicats et experts. La commission des affaires sociales a pris sa part. Nous avons déposé des amendements certains groupes par centaines que votre administration a enregistré, jour et nuit. Le renforcement des droits du Parlement est un combat que. Toujours mené à l'occasion de chacune des réformes constitutionnelles. Nous privons pas de ce droit d'examiner un texte fondamental comme des même il ne fait pas l'unanimité, c'est le principe de base de notre démocratie débattre. C'est ainsi le processus de. Bicamérisme améliorer pour avancer. Doit autant prendre le risque de reculer nécessaire et qui financier leur système de retraite. Car oui, le temps de la réforme est venue. Les chiffres ont été rappelés hier par mon collègue rapporteur le système sera déficitaire de 7 amené à hauteur de 1 milliard 800 millions d'euros le déficit pourrait atteindre plus de 13 milliards en 2030. La raison est simple, notre si régime de retraite et solidaire au point qu'il ne supporte pas l'allongement de l'espérance de vie. Il a le défaut de sa qualité. La solidarité intervient j'générationnel qui est au coeur de notre pacte républicain. J'ajouterai que le système par répartition est au coeur du pacte social.

Le RDS. A longtemps défendu une réforme systémique pour une retraite à points sa rancune. Face à l'abandon de ce projet. Hein tu as évoqué par le président de République mon groupe ne rejette pas en bloc votre projet. Monsieur le Ministre, qui au fond le fait qu'accélérer la réforme Touraine. Néanmoins, si nous sommes ouverts au compromis. Nous avons nous attendent. Les carrières longues le la. Revalorisation des droits des femmes, la compensation de l'engagement civique la pénibilité et l'emploi des seniors. Bien sûr. Et disons-le aussi, la participation de l'entreprise et il y a engagé des dividendes conséquents. En pleine crise du pouvoir d'achat ne doit pas être écartée. Il y a parfois de la naissance lorsqu'on le confronte le besoin de financement. Leur système de retraite et les chiffres des montants distribués aux actionnaires. Une réforme acceptable et à ce qui été partout doit reposer sur l'équité. C'est dans ce ça je dis nous faut travailler et à ne toutes les sensibilités ici bien sûr écoutez aussi nos concitoyens qui s'inquiète, mes chers collègues. Parce que le Sénat doit jouer son rôle, le RDS, je préfère le débat et si la grande majorité de mon groupe ne votera pas la motion référendaire. Merci monsieur le président. Je vais donner la parole. À notre collègue Alain Milon. Pour le groupe des Républicains. Vous la parole. La Suisse. Merci monsieur le président, monsieur le président. Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Madame la rapporteure générale. Mesdames et messieurs, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Déposer une motion référendaire. S'inscrirait dans une stratégie je cite à combattre sans obstrué. Stratégies ou stratagèmes. Nous sommes en droit de nous interroger. En effet. Les auteurs de la motion crie au scandale pour l'allongement de l'âge de la route de l'ouverture des droits à 64 ans en disant que l'on pousse les Français à travailler plus longtemps. Mais n'est-ce pas. Mes chers collègues, la réforme Touraine. Qui prévoit une durée de cotisation de 172 trimestres, soit 43 ans pour, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. la moyenne d'âge d'entrée sur le marché du travail et de 22 ans et si je compte bien à 22 plus 43 ça fait 65. Alors vous allez me répondre que les Français peuvent toujours partir à se passe de 32 ans. Oui mais avec quel retraite. N'ayant pas une retraite à taux plein leur pension subira une décote. C'est une machine en fait à créer des retraités plus pauvres et nous ne le voulons pas. Invoquer le référendum pour donner la parole au peuple sur un sujet qui le concerne directement témoignerait témoignerait. D'une volonté démocratique affirmé. Quel est le Synopsis. Mais qu'en est-il vraiment. Monsieur le Président Kader. Pourquoi déposer une motion référendaire dont les chances d'aboutir semblent bien minces. Pourquoi déposer une telle motion qui, si elle devait aller à son terme reviendrait à dessaisir le Parlement de son pouvoir de débattre de son pouvoir d'amender et donc de son pouvoir d'améliorer un texte particulièrement important en effet, à travers le prisme de la retraite. Nous parlons de travail. Nous parlons d'égalité homme femme. Nous parlons de justice sociale. Nous parlons de santé sujet qui m'est cher. Nous parlons de vieillissement. C'est donc un projet de société qui sous-tend ce texte et il serait illusoire. Hé bien naïf de penser qu'un référendum permettrait de répondre aux différents enjeux de la réforme des retraites. Au nom d'un retour à une légitimité populaire exprimée via un instrument de démocratie directe. La proposition de recourir au référendum revient à empêcher tout débat au fond. Pour être pertinent. Et exprimé une réelle volonté populaire. Le référendum d'apporter sur des questions claires précise concise et limiter. La complexité des situations liées à la retraite permettait de répondre à ces exigences. Ne risque-t-il pas de se muer en plébiscite, entraînant une personnalisation extrême du débat masquant les enjeux et cristallisant les tensions d'une société fracturée. Vous me permettrez de reprendre les propos du professeur Dominique Rousseau Dominique Rousseau qui lui- même a déjà été cité hier par notre collègue Éliane Assassi. Je cite Dominique Rousseau. La démocratie. A besoin d'institutions intermédiaires pour fonctionner sereinement et éviter une personnalisation excessive du pouvoir. Je cite encore le référendum laisse penser que ces institutions sont un obstacle à la démocratie. Alors quelles sont précisément les instruments qui font passer de la barbarie à la civilisation, C'est pourquoi je m'interroge. Sur cette volonté de s'auto-mutiler. Après des débats affligeant à l'Assemblée nationale, tout le monde l'a dit qui ont encore davantage assombri d'image des parlementaires et creuser le fossé entre élus et citoyens. Il est particulièrement important. Voire vital pour la démocratie représentative d'assumer notre mission d'exprimer clairement nos positions et de défendre nos opinions. Les syndicats ont, de ce point de vue jusqu'à ce jour, fait preuve de responsabilité en jouant leur rôle. Les élus politiques seraient-ils moins incapables que les élus professionnels de remplir les obligations de leur mandat. Je pose la question, J'espère et je suis persuadé. Que tous ensemble dans cet hémicycle, nous saurons avec détermination conviction faire évoluer ce texte, Monsieur le Ministre, cette réforme n'est peut-être pas proposer au bon moment. Il aurait fallu que le gouvernement prenne en compte les propositions du Sénat beaucoup plus tôt. 2019, depuis 2019, la commission des affaires du. Des affaires sociales du Sénat, recommande l'adoption de la réforme paramétrique des retraites afin de préserver la soutenabilité financière du système et donc sa pérennité, pour les générations futures. Serge René-Paul. Nous devons agir pour ne pas laisser filer les déficits. Je vous rappelle, plus de 150 milliards d'euros cumulés. Pour les 10 prochaines années. Et ces prévisions sont très optimistes puisque basé sur un taux de chômage à 4,5%. Cette réforme est donc urgente. Proposée par la majorité sénatoriale depuis plusieurs années le report de l'âge légal et l'allongement de la durée de cotisation vont enfin être mises en oeuvre. Mais si nous partageons la philosophie globale du projet pour garantir la pérennité de notre système, nous avons fait de nombreuses propositions pour améliorer la situation des Françaises et des Français, en particulier celle des seniors, celle des mères de famille, celle des enfants orphelins et celle du handicap il faudra relire le texte vous vous réveillerez que c'est vrai. Si vous dit c'est pas vrai c'est parce que vous n'avez pas lu. Nous souhaitons également promouvoir un système plus équitable, notamment à travers la lutte contre la fraude et la participation de tous les salariés à l'effort de travailler plus. Nous aurons l'occasion, mes chers collègues d'y revenir en détail au cours de l'examen des articles et des discussions. Mes chers collègues, nous ne pouvons renoncer à nous prononcer sur ce texte. Nous ne pouvons pas nous défausser. C'est pour toutes ces raisons que le groupe LR ne votera pas cette motion et que nous consacrerons le temps imparti à un débat argumenté. On nous appuyant sur le travail considérable. Réalisé par nos rapporteurs. Je vous remercie. La parole est maintenant notre collègue Daniel Chassain. Pour le groupe les indépendants. République et Territoires. Monsieur Chassaing vous avez. Monsieur le président. Monsieur le ministre. Madame la présidente de la commission, mesdames, messieurs, le rapporteur. Mes chers collègues. Le programme du président de la République, candidat avait dans son programme le départ à la retraite à 64 ans mais c'est vrai que beaucoup ont voté pour faire opposition au RN. Le Sénat. A aussi depuis plusieurs années. Voter un amendement. Concernant cette mesure d'âge au PLFSS pour le départ en retraite. Mais mes chers collègues, si les comptes de la branche retraite était en voie de l'amélioration. Il serait je pense agréable à tous de renoncer à ce projet. Qui mobilise c'est vrai les syndicats que j'ai rencontré dans mon département et beaucoup de Français hostiles à cette réforme. Nous savons tous que la branche retraite va se dégrader cela est confirmé par le corps avec ça vient d'être dit par Alain Millon. millions milliards par an en 2030, 26 en 2040. Pourquoi. Bien je répète ce que j'ai quand même dit hier mais je le répète, le nombre de cotisants pour un retraité passé de 4 en 1970 à 2 en 2001,7 En 2000, en 1970, l'espérance de vie était 70 ans pour les hommes et 76 pour les femmes, on est passé à 79 et 86, nous étions. À ce moment-là 4 millions de retraités. On est à 17 millions et 21 en 2030. les générations futures risquent de ne plus pouvoir assumer les de retraite par répartition, mis en place en 1945. Si des cotisations doit augmenter pour maintenir le pouvoir d'achat des retraités. D'autre part, ça a été dit, le dynamisme démographique qui a été longtemps une forte de la France des croix. Les faits sont là, et nous devons débattent pour équilibrer les retraites sans majorer les cotisations en augmentant le travail le plus légèrement possible afin de maintenir les retraites parti à répartition et la sécurité sociale. C'est pour cela que j'avais souhaité une loi travail. Avec une concertation avec les partenaires sociaux avant ce projet de loi. Cela afin que les personnes handicapées invalides carrières longues les femmes puissent avoir une retraite plus tôt mais aussi une meilleure prise en compte des critères de pénibilité. Tout ça avec les partenaires sociaux renforcer les trimestres. Travaillé pour les enfants. Renforcer les les employes seniors cumul emploi-retraite avec de nouveaux droits pour les aidants pour la revalorisation des petites retraites intégration de l'apprentissage a ça de de trimestres etc valoriser également les engagements au niveau associatif et bien d'autres pour lesquels, mes chers collègues, vous avez fait des amendements sur ce texte. Cela bien sûr me semble être de la compétence des affaires sociales du Sénat. D'autre part. J'avais fait un amendement j'ai fait un amendement de revoyure en 2027 afin de faire un bilan et pourquoi pas rajouter en fonction des résultats, hé bien un autre moyen de financement. Et si amélioration mais pourquoi pas faire marche arrière mais ça se m'étonnerait. Mais pour en revenir au référendum quelle question allez vous poser la question sur le recul de l'âge légal sûrement mais aussi est-ce que vous allez poser la question de la suppression de la loi Touraine mises en place sur le quinquennat de François Hollande avec 172 trimestres. 43 ans de cotisation pour une retraite complète. que si cette loi Touraine et conserver en l'état pour 43 ans de cotisation 2035 hé bien pour une personne née en 1900, société enterrons ce qui a débuté son travail en 1992 à 21 ans, il partira avec une retraite à taux plein. 43 ans plus tard, c'est-à-dire en 2035 mais il aura 64 ans. Est-ce que François Hollande a fait ça pour brimer les Français mais non c'est bien pour équilibrer les retraites. Les Français savent bien qu'une réforme ne peut pas se résumer à une simple question fermée sur autant de projets essentiels, cité Il est donc nécessaire d'avoir un véritable débat démocratique, c'est au Sénat que nous pouvons amender ce texte pour mieux tenir compte des situations particulières. Par ailleurs, je rappelle que aucun des précédents projets de réforme des retraites n'a déjà passé par un référendum, nous c'est donc donc débattre amender ce texte pour une réforme la plus juste possible. Le groupe les indépendants rejettera cette motion de référendum. Merci, bonsoir. Donner

Merci monsieur le président, Monsieur. Monsieur le Ministre Mesdames et messieurs les d'amener les rapporteurs. L'examen d'une motion référendaire. Une première dans cette enceinte depuis une décennie est un moment d'une extrême gravité démocratique. Nous parlementaires n'avons pas vocation à nous dessaisir de la mission que nous ont confié les citoyennes et les citoyens de délibérer et voter la loi. Et si nous sommes favorables à davantage d'implication citoyenne dans la fabrique de la loi, la binarité du référendum sommes souvent peu compatible avec l'exercice complexe de rédaction et de vote de la loi. Alors pourquoi cette motion. Tout d'abord parce que ce débat parlementaire est une farce. Le gouvernement a choisi un véhicule législatif inadaptée jamais utilisé pour une réforme de cette ampleur qui Corse cette. Le débat dans le temps et dans l'espace en interdisant de l'élargir au-delà des paramètres financiers symbole s'il en est que pour vous le nez travail n'est qu'un coup. Au moins en son temps, Édouard Philippe avait eu le courage de proposer un vrai projet de loi et une vision nous la confession évidemment mais elle avait le mérite de proposer autre chose, autre chose qu'une réforme de comptable en costume gris destiné à faire payer aux travailleurs les cadeaux fiscaux offerts aux entreprises et aux plus aisés. Le Sénat doit donc examiner et c'est une délétère. Première historique, un texte qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale qui doit absolument être voté avant le 12 mars minuit, faute de quoi le carrosse redeviendra citrouille. Mais et nous sommes ici en absurdie la citrouille peut tout de même faire l'objet d'un examen en commission mixte paritaire ou d'une adoption par ordonnance. La 5ème République n'est jamais en reste pour piétiner le Parlement mais la présidence Macron à innover comme aucun autre avant. Dans la dérive autocratique d'un exécutif hors-sol isolée dans sa tour d'ivoire isolé ou devrais-je dire plutôt dire assiégée. Non content de mépriser le Parlement de mépriser les partenaires sociaux de lever contre vous un front social qui comme rarement c'est qui comme rarement. C'est le peuple de France tout entier que vous méprisez. Depuis des mois, tous les sondages affichent une opposition ferme et constante oscillant entre 2 tiers et les 3 quarts de nos concitoyens. Plus vous méprisez leur Intelligence et invoqué le besoin de faire de la pédagogie de votre réforme, plus les Français s'y opposent les manifestations enregistre, semaine après semaine des records de participation et les préavis de grève tombent les uns après les autres pour faire du 7 mars et de la prochaine semaine un moment historique de l'histoire du mouvement social. Alors que nous sortons à peine de la pandémie, alors que la guerre gronde aux frontières orientales de l'Europe alors que l'inflation explose, alors que la crise climatique nous heurte plus fort que jamais au point de nous obliger à rationner l'eau source de toute vie. Vous n'avez aucun scrupule à conduire le pays tout entier au blocage. Mais pour quel besoin, pour qu'il y urgence est la nécessité d'un agenda caché de vos négociations avec la Commission européenne ou est-ce la seule fierté mal placée du président de la République, il considère que le barrage à l'extrême droite vaut adoubement de sa royale personne et qui n'a même pas pris la peine d'étudier la composition de la potion qu'il entend faire boire au pays et à laquelle il n'a visiblement pas compris grand chose. Le retrait de ces textes s'impose cependant pour vous éviter de perdre la face, nous vous proposons une solution alternative. Soumettre donc ce projet dont vous êtes si fier à l'approbation des Françaises et des Français, ils sont 70% à le demander 70% à vouloir se prononcer sur cette réforme, 70% à vouloir être maîtres de leur propre destin 70% à vouloir exprimer leur parfaite compréhension de votre projet de ces prétendues mesures de justice, d'égalité, femmes-hommes et de prise en compte de la pénibilité. Tout à sa réélection, dont il ne cesse de se prévaloir abusivement Emmanuel Macron alors interrogé sur la possibilité d'avoir recours au référendum sur la réforme des retraites. Déclaré le 11 avril. Je n'exclus pas le référendum pour quelque forme que ce soit, je l'ai dit, je suis pour le retrouver notre discussion ne permet de clarifier les choses. L'occasion est ici toute trouvée ce même Emmanuel Macron qui en a appelé au bon sens des Français à l'occasion de leur faire réellement confiance. Mes chers collègues. Notre démocratie est malade il est inconcevable de trouver dans nos, dans nos deux chambres, une nette majorité pour progrès j'ai rejeté par la grande majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens notre représentativité et dramatique et d'autre légitimité légitimité Il convient, une fois n'est pas coutume de nous dessaisir de cette réforme, de ne pas voter brutalement dans un déni de démocratie manifestent cette réforme bricolée dont personne ne veut. Nous avons besoin, comme le disait De Gaulle, de savoir ce qu'il en est dans les esprits et dans les coeurs. Mes chers collègues de droite soyez gaulliste n'ayez pas peur du peuple voter cette motion référendaire. J'ai donné la parole à notre collègue. Ali le héros pour le groupe socialiste. Écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre, madame la présidente madame la rapporteure, chers collègues. Dans un entretien au Monde l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon souligne que si le président de la République peut se prévaloir d'une légitimité procédurale née de son élection, il lui manque la légitimité sociale fondée sur l'intérêt général et la perception citoyenne. Nombreux sont les Français et les Françaises qui ont utilisé le bulletin de de votre de vote Macron pour faire barrage à l'extrême droite mais pas pour soutenir sa réforme des retraites. Le président de la République ne peut se prévaloir d'une légitimité pour faire cette réforme, alors même que la France se soulève, quel sera à l'arrêt, le mardi 7 mars pour dire son opposition. Cela a été rappelé notre système de retraite, elle l'héritage de combat et de conquêtes sociales passées. Rien ne justifie une telle obstination. Renforcé par la droite sénatoriale, notre système actuel est excédentaire en 2022 et son évolution et contrôlé le rapport du conseil d'orientation des retraites de l'firme il n'y a ni urgence ni nécessité le déficit se résorbera grâce aux réformes entreprises pour stabiliser la part des retraites dans notre PIB. Il n'y a pas de dérapage des dépenses, il y a nécessité d'ajuster nos recettes. Nous avons des propositions réalistes pour un ajustement soutenable et équitable sans imposer 2 ans de travail obligatoire pour toutes et tous. La mobilisation inédite des Français et des Françaises. Pour exprimer avec force et détermination. Qui ne veulent pas travailler 2 années de plus alors que les conditions de travail les rendent incapables de poursuivre leur activité. Votre réforme ne fait que des perdants. Certains plus que d'autres et les plus touchées sont les catégories populaires et les femmes. Le président de la République déclarait lui-même pendant la campagne présidentielle de 2017 je cite après plus de 20 ans de réformes successives, le problème des retraites n'est plus un problème financier. Alors voilà qu'aujourd'hui l'urgence financière justifie votre choix de procédure PLFSS rectificatif. Venons-en donc à la forme tous les Français sont concernés par les retraites. Vous affirmez que le président Zidan a été élu en connaissance de cette réforme vous vous omettez de rappeler que le 3ème tour des élections nationales directe de 2022 ne vous a pas donner une majorité solide à l'Assemblée nationale pour la mener à bien et nous avons ici au Sénat, un texte qui n'a pas été soumis au vote de l'Assemblée nationale. En restreignant le temps des débats au Parlement en utilisant l'article 47. 1 de la Constitution. Vous avez vous même créé là les conditions de l'obstruction, comment pouvez vous considérez la réforme des retraites comme une simple rectification budgétaire qui n'impacte d'ailleurs que faiblement l'année 2023, alors que vous privés des 2 meilleures années de leur retraite. L'usage de cette procédure d'urgence et le contenu de la loi est contestée par le Conseil d'État et le sera bientôt par le Conseil constitutionnel face à l'incapacité du gouvernement de faire voter ce texte. Dans les 2 chambres, soyez à l'écoute de l'opposition du peuple. Je vous appelle à voter cette motion référendaire en vertu de l'article 11 de la Constitution pour que le peuple tranche. Un référendum sur un sujet aussi essentiel que celui des retraites permettrait au gouvernement de vérifier l'adhésion ou pas du peuple français et à monsieur Macron de vérifier son postulat d'accord tacite des Français sur la réforme les Français et les Françaises veulent prendre leur retraite de leur vivant, nous la soutenons avec force, vous l'aurez compris, notre groupe socialiste, écologiste et républicain. Soutiendra cette motion référendaire pour associer le peuple français à cette réforme de société, et je vous invite à droite à vous associer en votant pour cette motion à vous remettre au peuple ça légitime a tranché nos débats dans le contexte de rejet qui s'exprime dans la rue avec une unité syndicale

merci monsieur le président, madame la présidente de la de la commission mais madame et messieurs, monsieur le rapporteur. Quelques mots pour dire qu'évidemment et. Et sans surprise, le Gouvernement est défavorable à l'adoption de la motion référendaire qui a été proposé. J'ai entendu finalement 3 arguments ou 3 questions auxquelles je souhaite apporter les les positions du gouvernement en réponse première argument concerne. La question de la recevabilité. Nous avons évoqué ce sujet hier, est-ce que cette réforme doit être porté dans le cadre d'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif. Nous avons eu l'occasion hier. La rapporteure générale moi même d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse et de rappeler que le cadre dans lequel nous sommes. Les conséquences de cette réforme sur les comptes sociaux pour l'année 2023 rendent à la fois légitime recevable et donc justifier le recours à un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Il y a malgré tout et c'est une parenthèse que je fais quelque chose d'assez cocasse, pardon pour cette expression à entendre reprocher au gouvernement d'avoir organisé une forme de d'obstruction pour 2 raisons, la première c'est que le, le temps de débat dont dispose le Parlement sur cette réforme est supérieur. Autant de débats dont a disposé le Parlement sur les deux réformes précédentes et les choix faits par le Sénat d'ouvrir un nombre de jours supplémentaires par rapport à l'Assemblée nationale vient illustrer ou conforter celui-ci puis il y a une 2ème raison c'est que, à ma connaissance ce n'est pas le gouvernement qui, devant l'Assemblée nationale a déposé plus de 20.000 amendements, dont des séries identique. Je peux vous assurer que j'avais plus ah d'entrer dans le sujet de fond que d'examiner ces amendements identiques. La, la 2ème. Question à laquelle je veux apporter la position du gouvernement. Concernent finalement la la légitimité ou l'intérêt qu'il y a à. Maintenir au Parlement. Cette capacité à apporter examiner la la réforme des retraites. Et à, à travailler sur ces questions là, je crois très fortement à cette l'Égypte légitimité de la démocratie représentative et du parlement pour débattre des retraites. J'y crois parce que l'histoire récente nous a montré. Que toutes les réformes des retraites depuis 1980

Mais le le Parlement toujours saisi de cette question des retraites et a pu accompagner, mettre en oeuvre des, des progrès qui sont des progrès très substantiels pour l'ensemble des assurés. Je ne prends qu'un exemple qui a été évoquée, notamment par. Le président et qui est, c'est la question des carrières longues. Lorsque l'on se retourne sur un passé récent. À 20 ans. Avant 2003. La l'âge de départ à la retraite était de 60 ans la durée de cotisation requise était de 37 ans et demi et dans un système tels que on le connaissait un assuré une assurés qui travaillent qui faisait des études une licence, une maîtrise qui entrée sur le marché du travail à 22 ans et demi travailler très exactement 37 ans et demi et bénéficier d'une retraite à taux plein à 60 ans et dans le même temps. Ses camarades de classe à l'école. Vous pouvez commencer à travailler très tôt à 14 ans à 15 ans la saison et devait aller jusqu'à 60 ans et ainsi cotiser 44, 45 46 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein, c'est la création du dispositif de carrières longues dans la réforme de 2003 qui a apporté une première réponse et depuis chaque réforme, examinée, débattue et adoptée par le Parlement, a permis de diminuer cet écart de durée de cotisation à l'échelle d'une vie pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous arrivions à une situation et ce sera encore plus vrai. Cette réforme est adoptée, où l'écart de durée de cotisation requise sera finalement ramené à à moins d'un an parfois à quelques trimestres parce qu'on sait qu'il n'y a pas de de perfection en la matière et ce seul exemple montre qu'il y a un intérêt à ce que le Parlement puisse se saisir ces sujets les creuser les amender les approfondir et des dispositions techniques qu'un examen par voie référendaire ne permettrait pas. Enfin. La 3ème. Question à laquelle je veux apporter une réponse c'est justement quel serait l'intérêt, quel serait l'utilité ou l'opportunité plutôt de la démarche de confier cette question ce ce débat et cette réforme a une question référendaire je crois et ça a été dit par plusieurs intervenants que la complexité du sujet, je l'évoquais hier en réponse à la discussion générale a interdit cette démarche interdit cette démarche parce que aucune réponse binaire ne peut constituer une réponse à la question des retraites. Il a été évoqué par plusieurs intervenants et avec des angles très différents. La la question des femmes et en particulier la question des mères puisque ont été évoquées les questions relatives au trimestre accordés et validé à l'occasion d'une maternité ou au-delà des trimestres accordés pour l'éducation des enfants. Je, je suis convaincu, mais ça peut faire l'objet d'un débat. Je suis absolument convaincu que pas un couple. Aucun parent. Aucune femme ne décide d'avoir un enfant pour espérer avoir en contrepartie. Telle ou telle trimestres telle ou telle majoration, c'est un projet de vie, c'est un projet personnel. C'est une construction par contre je suis absolument convaincu. Que la maternité, tout comme le fait d'élever des enfants. Peut être soit un frein à avoir un empêchement à cotiser soit un frein à la progression à la promotion professionnelle et donc un facteur d'inégalité professionnelle. Le système de retraite ne ne compte rien, aucune disposition qui soit de nature à marquer crée une inégalité entre les femmes et les hommes. Il traduit-il retranscrites dans le calcul des pensions. Non pas une volonté d'inégalités mais l'accumulation d'inégalités tout au long de la vie et c'est évidemment la question de l'égalité professionnelle qui apportera la seule et vraie réponse soutenable à la question de l'égalité des pensions entre les femmes et les hommes. Par contre notre système ne doit pas s'empêcher de réparer. Et c'est pour ça que j'ai dit hier. Combien. Regardons avec bienveillance l'amendement proposé par le président Retailleau adopté par la commission des affaires sociales. Pourquoi. Parce que d'une part il permettra. Il permet. De de maintenir un système, un système qui autorise une femme je parle uniquement des trimestres liées à la maternité. Les 4 dans le régime général, les deux dans le secteur public et cela renvoie au débat sur les droits familiaux que j'évoquais permettra à des femmes ayant des carrières hachées. De pouvoir grâce à ses trimestres validés compléter leur carrière éviter la décote. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est pour ça que trimestres ont été pensés dans un, dans un 1er temps, qu'on ne me des contreparties et des trimestres qui ne pouvait être cotisés au moment. De la grossesse et de l'accouchement et dans un 2ème temps quand même un, un une réponse peut être au aux carrières mais nous avons une situation qui fait qu'avec l'augmentation pas celle-ci mais l'augmentation depuis. 1993 depuis 2003. Pardonnez-moi de, de l'âge de départ à la retraite. Nous avons une situation ses trimestres dit de maternité. Peuvent dans certains cas dans le cas où les femmes ont une carrière complète au quasiment complète perdre d'une certaine manière le leur utilité. Dès lors, ou que la carrière peut être complète sans avoir recours aux besoins de ses trimestres. Et dans ce cas-là il faut se demander quelle est l'utilité de ces trimestres et l'utilité de ces trimestres peut être non pas de compenser une incapacité à cotiser pendant un temps mais à compenser les inégalités de carrière que peuvent encore. Provoquer susciter et malheureusement le fait d'avoir des enfants et et de consacrer du temps à leur éducation et donc l'alternative qui est ainsi proposé à la fois maintenir ce bénéfice de temps pour les femmes qui en ont besoin du fait d'une carrière hachée mais permettre à celles qui ont une carrière complète ou quasiment complète quelques trimestres avant l'âge d'ouverture des droits, de bénéficier d'une surcote parce que finalement. La démonstration est peut-être un peu simpliste. Si elles ont réussi à avoir une carrière complète. Cela signifie que leur grossesse, leur maternité ne les a pas empêchés de mener une carrière mais peut les avoir empêchés de progresser aussi rapidement que leurs collègues hommes et donc permettre à ces femmes qui ont une carrière complète au quasiment complète à l'heure de ne bénéficier non pas de temps validé mais d'une surcote en terme de pensions nous paraît permettre une alternative intéressante et posant une première Pierre, une première brique pour le chantier des droits familiaux que nous aurons à aborder et élaborer d'ici le PLFSS 2024 j'ai pris cet exemple qui renvoie là encore à la complexité que j'évoquais hier pour dire tout simplement et j'en termine par là qu'une question binaire à laquelle on apporte une réponse par oui ou par non, est une question trop simple, trop Direct et donc inopportune pour aborder une réforme comme celle-ci je compte plus sur la richesse des débats du Parlement pour permettre d'améliorer le texte. La discussion générale est donc Close. Nous allons passer aux explications de vote sur la motion. J'ai donc j'ai déjà de demandes d'explications de vote. Monsieur de notre collègue Breuiller.

Mais bien sûr aussi. Nous vivons une crise démocratique d'une grande profondeur tant l'écart entre le peuple et le gouvernement ne cesse de s'accroître. Étant l'écart entre l'immense majorité de nos concitoyens et la majorité de notre chambre et grand. Des millions de personnes manifestent le sentiment d'injustice sociale et d'une profondeur rarement atteint l'Unit l'unanimité syndicale s'exprime face à cette réforme. Et chers collègues, si nous ne bougeons rien le populisme sans nourrira. Alors comment sortir de cette crise démocratique. Nos collègues du groupe centriste appelle à l'ouverture d'un grand débat social. C'est une position que je trouve pour ma part très intéressante et très intelligente tente on ne peut pas parler des retraites sans parler du travail lui-même ce que ce texte ne permet pas parce qu'il est inscrit dans un texte rectificatif de finance. Mais cette proposition de nos collègues centristes suppose une seule chose. C'est que le débat commence par ce round social. Et pas par le vote d'une loi. Ici, nous faisons tout à l'envers. Sous l'impulsion de ce gouvernement nous changeons le mix énergétique avant le débat sur les choix énergétiques et nous votons une réforme de la retraite avant le débat sur les sujets du travail, c'est un problème démocratique qui nourrira des populistes. Des citoyens appellent à une convention. Ah une Convention citoyenne sur ce sujet des retraites, moi j'avoue que cette idée me séduit parce que je m'étonne jeune sénateur qu'en aucun cas nous ne parvenons ici à trouver des consensus et que lorsqu'on réunit des conventions citoyennes sur des sujets aussi délicats que la fin de vie ou le climat, ils soient capables d'élaborer ces consensus, il y a là un problème qui doit nous faire réfléchir nous parlementaires sur cette façon dont le débat est finalement bloqués à l'intérieur de nos institutions. Alors il reste la dernière proposition, celle du référendum. Elle a de graves inconvénients notamment par son côté binaire. Mais il n'y a jamais de honte à redonner au peuple, la capacité de décider. Mes chers collègues, après chaque élection. On découvre un taux d'abstention abyssale. Fait des grandes déclarations sur la crise démocratique. Et puis à peine le temps passant, on finit par oublier la gravité du décrochage d'une large partie de notre population notamment dans le monde salarié avec les choix politiques du pays. Et la, et pourquoi. Parce que depuis des années et des années. Sont voter des réformes qui comme un rouleau compresseur attaquent notre modèle social et notre modèle républicain. Et on ne peut jamais rien. Au vote, on fait l'alternance ça change pas beaucoup. On vote pour un président qui nous dit bah mon programme, tout mon programme, alors qu'il s'est fait élire contre Marine Le Pen. Les gens n'y croient plus à cette démocratie. Il est donc fondamental de retrouver un nouvel équilibre entre le choix référendaire qui donne au peuple la parole ou en général il vote. Et de l'autre côté la démocratie représentative. Si on n'avance pas sur les 2 jambes. Les deux vont être affaibli. Or là, de quoi s'agit-il. Il s'agit pas de sous tailles. On peut toujours faire des amendements un PLFSS pour améliorer la condition de la retraite des femmes et ceci ou cela. C'est l'essentiel. Le référendum doit avoir lieu sur l'essentiel, c'est-à-dire le recul de l'âge de la retraite légal à 64 ans que massivement notre pays refuse. Et ne pas vouloir faire ça s'est creusé la tombe de nos de notre vision républicaine s'est creusé la tombe de notre démocratie. Alors mes amis. De air mes amis, mes collègues mais néanmoins amis de LR. Je vous rappelle non seulement le général de Gaulle. Mais comment c'est pas à nous raconter que le référendum n'est pas une bonne chose parce que pour pour faire un référendum sur l'immigration. Alors ça madame Pécresse tombe tambours et trompettes.

Merci monsieur le président. Alors, le constat est sans appel, l'IFOP, 75% des ouvriers employés 63% des quads sont opposés à la réforme. 59% sont favorables à une augmentation des cotisations Elabe, 77% des actifs jugent la réforme injuste 66% inefficace 61% pas nécessaire. 72% des actifs soutiennent la mobilisation et 60% souhaitent qu'elle se durcisse avec des blocages. Aussi 59% trouvent que le responsable du conflit social et déblocage et le gouvernement. Toutes ces enquêtes ne font que mettre au grand jour l'opposition massive et sans équivoque de la population et des actifs qui trouvent eux aussi que le retrait est non négociable. La démocratie c'est le régime du peuple pour le peuple par le peuple et pourtant vous nier la légitimité sociale de la population et des syndicats majoritairement opposés au projet Rosanvallon complète Rousseau chers collègues millions et ce pour la seule légitimité électorale, d'avoir été élu alors que chacun sait que vous le devait d'abord aux circonstances du second tour n'était pas un blanc-seing à votre programme et certainement pas. À ce prolongement de de l'âge de la retraite. Vous faites semblant aujourd'hui de l'oublier, vous le disiez entre les 2 tours pour demander nos voix. La population doit avoir le droit de débattent et cette réforme de de cette réforme et retrouver la parole alors que vous beaucoup tronquée aujourd'hui le débat parlementaire. Si le peuple vote contre la réforme du gouvernement. Il ne vous restera que le retrait ou de dissoudre le peuple comme disait Bertolt Brecht. Les écologistes, donc pour toutes ces raisons soutiennent cette motion référendaire. Si. Monsieur le président, mes chers collègues, je voudrais simplement vous rappeler que le référendum, le référendum est un outil, un outil démocratique qui permet de trancher. Dans un moment de doute un certain nombre de questions et il me semble que nous sommes au coeur. De ce doute. Et je pense donc que le référendum est nécessaire. Alors. Bien évidemment il y a des réticences du président de la République il y a des réticences du du gouvernement pour convoquer un référendum mais je dois dire que ça ne m'étonne guère car ce qu'ils craignent. Et un peu ce que craignent aussi nos collègues de la majorité sénatoriale ce qu'ils craignent c'est une remise en cause de leur légitimité. Or ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout le sujet. Et si monsieur Macron se félicite et cela a été dit du bon sens des Français. Il doit aller donc au bout de sa logique et favoriser l'expression de ce bon sens et non la crainte. Je pense que rejeter cette motion, c'est envoyer. Un message très mauvais au au 90% d'actif et au soir plus de 60% de Français qui veulent le retrait de ce texte parmi lesquels je voudrais insister, parmi lesquels des électrices et des électeurs de Macron au 1er tour de la présidentielle, mais aussi des et électrices et des électeurs qui soutiennent et ont voté pour les candidates et candidats de la droite, qu'elle soit LR ou centristes aux dernières élections, on peut s'interroger sur leur niveau de tolérance de ces électrices et ses Lecteurs car cette réforme vient compléter des contraintes financières et sociales qui leur sont imposées depuis plusieurs années maintenant, donc la colère et la le ressentiment et là il serait temps que vous sortiez de votre bulle pour entendre non seulement les flatteur, mais surtout en temps de celles et ceux qui. Et exige pardon le retrait de ce texte. Pour notre part et nous en sommes signataires, nous soutenons cette motion référendaire. Monsieur Jomier pour quatre Cameron. Merci. Monsieur le président. Quand on en arrive dans nos débats a invoqué le général de Gaulle je sais en général qui a un grand trouble au fond dans l'assemblée. il y a un grand trouble et un désordre institutionnel et il ne date pas des débats à l'Assemblée nationale et de comportement. Les comportements auxquels on a assisté, il vient de bien plus loin ce désordre institutionnel. C'est le chef de l'État qui en est responsable. Car dès son 1er mandat il a marqué son mépris des organisations intermédiaires. Il a quasiment théorisé même et ce mépris des organisations intermédiaires. Il s'est déroulé et aujourd'hui il explose à la figure du Parlement. Pour contourner les organisations. Parce qu'on peut. On peut mener une réforme de retraites en négociant et en ayant au moins la sentiment d'une partie des organisations syndicales, ça n'est pas si ancien dans notre histoire, je vous le rappelle mais c'est pas le Paris qui a été pris par le chef de l'État, c'est de les contourner. Résultat, un front syndical total, remarquez ce gouvernement nous y habitue avec les professions de santé, c'est la même chose. Il arrive à tous les ligués contre lui et a échoué à signer un accord conventionnel, je ferme la parenthèse mais ça n'est pas une parenthèse, c'est sa ligne de conduite et donc il arrive au Parlement et face à un peuple qui dit non. Face à des organisations syndicales qui disent non, il imagine une procédure institutionnelle qui est bancal sur le plan constitutionnel et qui met le Sénat dans la situation d'être l'Assemblée du peuple, ce que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas, nous sommes la chambre des territoires. Eh bien c'est un désordre institutionnel total qu'a créé le chef de l'État c'est un chaos qui ne peut pas se résoudre de façon apaisée par la voie parlementaire et croyez bien que je le regrette. Il n'y a qu'une solution c'est de retirer ce projet. Hé oui c'est d'aller vers le peuple.

J'ai entendu dans les arguments s'opposant à cette motion référendaire des. Plaidoyer pour la démocratie parlementaire. Je prends date parce que oui le Parlement. Oui l'Assemblée oui le Sénat. c'est le fondement du fonctionnement démocratique dans notre République. Et donc. Très souvent, on a dû le défendre quand il a été brutalisé par différents gouvernements et en particulier depuis Emmanuel Macron cette brutalisation est constante depuis. Quelques années les procédures d'urgence. Qui devait être. Exceptionnel sont la règle sur la coutume. Donc, mes chers collègues qui venait faire ses plaidoyers. Et Monsieur le Ministre, en particulier. Pourquoi à chaque fois à ce point le brutaliser. Mais on est dans une situation très particulière. On ne va toucher à la vie de millions de nos concitoyens. Alors que le président de la République. Dans son élection. N'a pas été investi par le peuple de faire cette réforme et d'ailleurs s'il avait été, ça se serait vu aux législatives il aurait une majorité. Et donc on est devant une réforme majeure qui touche à la vie de millions de nos concitoyens. Et le message et le mandat parlementaire n'est pas clair. Celui du président, celui de la Première ministre, celui des majorités. Et en plus de cela. Une mobilisation syndicale qui est massive. Et des enquêtes d'opinion qui tousse. Disent qu'une grande majorité de Français contre et donc la seule façon de dénouer cette crise. Cette crise démocratique sur cette question et que le peuple prenne la parole par voie référendaire. Et ça veut dire un débat dans le pays bien entendu. D'autres demandes d'explications de vote. Je n'en vois point. La discussion. Donc nous allons passer. Au moment du vote sur l'article unique de la motion de renvoi au référendum. Je rappelle qu'en application de l'article 59 du règlement de scrutin public et de droit. Donc. C'est l'article 56 du règlement qui est appliqué, maintenant le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter.

Le scrutin est clos.

En conséquence, mes chers collègues. Nous allons poursuivre la discussion du projet de loi de financement. Projet de loi. Rectificatif de la Sécurité sociale. Je vais maintenant suspende la séance elle sera reprise à 17h pour l'examen des Arctic la séance est suspendue. Je souhaite bon courage à la commission. La séance est suspendue.